Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses, dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je rappelle que l'auteur de la demande dispose d'un temps de parole de huit minutes, puis que le Gouvernement répond pour une durée équivalente.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les violences sexuelles sur mineurs constituent une réalité insupportable, voire difficilement concevable pour beaucoup d'entre nous comment imaginer que les êtres les plus vulnérables et les plus innocents dans notre société puissent être victimes de telles agressions ? Celles-ci sont pourtant beaucoup plus fréquentes qu'on ne l'imagine. Si elles se produisent majoritairement dans le cadre familial, elles peuvent aussi être commises par les adultes qui prennent en charge les mineurs dans un cadre professionnel ou associatif. C'est à cette seconde catégorie de violences sexuelles sur mineurs que la mission commune d'information que j'ai eu l'honneur de présider a consacré ses travaux. Ils ont abouti à l'adoption d'un rapport d'information le 28 mai dernier. Ce sont d'abord les abus sexuels révélés au sein de l'Église catholique qui ont conduit le Sénat à s'intéresser à ce sujet. Nos collègues du groupe socialiste et républicain, que je remercie de leur initiative, avaient demandé la constitution d'une commission d'enquête qui aurait travaillé spécifiquement sur ce sujet. Le bureau du Sénat a jugé préférable de retenir un champ d'investigation plus large, afin d'examiner comment la prévention, la détection, le signalement et la répression des infractions sexuelles sur mineurs sont organisés dans les différentes structures qui accueillent des enfants et des adolescents, qu'il s'agisse de l'éducation nationale, des associations sportives, des services de l'aide sociale à l'enfance, des services de garde d'enfants, des associations sportives, des établissements d'enseignement culturel et artistique, des colonies de vacances et des centres aérés. Pour dresser ce panorama, la mission a procédé à une cinquantaine d'auditions, complétées par trois déplacements. Ce travail n'aurait pas été possible sans l'investissement et la disponibilité de nos trois rapporteures, que je salue : Marie Mercier, qui a déjà eu l'occasion de travailler sur le droit pénal applicable aux infractions sexuelles sur mineurs, Michelle Meunier, qui connaît très bien les politiques de protection de l'enfance, et Dominique Vérien, qui a notamment approfondi la question de la prise en charge des auteurs de violences sexuelles sur mineurs. Le rapport d'information formule trente-huit propositions, que nous aurons l'occasion d'évoquer au cours de ce débat. Nous avons bien sûr travaillé en ayant toujours en tête l'intérêt des victimes. Comment favoriser la libération de la parole, indispensable pour que les faits soient connus et sanctionnés ? Comment les aider à surmonter le traumatisme de l'agression ? Surtout, comment éviter d'avoir à déplorer de nouvelles victimes, ce qui pose la question de la prévention de la récidive et de la prévention du premier passage à l'acte Nous avons constaté, dès le début de nos travaux, qu'il existait peu de données précises et actualisées concernant le nombre de victimes et le contexte dans lequel surviennent les agressions. Cela nous a conduits à recommander la mise en place d'un observatoire, partant du principe que l'on ne peut combattre efficacement que ce que l'on connaît bien. Nous avons également constaté que les pratiques et les règles en vigueur variaient beaucoup d'un secteur à l'autre les contrôles sont par exemple systématiques et automatisés pour tout ce qui concerne les accueils collectifs de mineurs- c'est-à-dire les colonies de vacances et les centres aérés ils paraissent en revanche plus aléatoires dans le monde du sport, alors que nous savons que la relation de proximité qui s'établit entre un entraîneur et un jeune athlète peut favoriser l'apparition de phénomènes d'emprise pouvant déboucher sur des agressions. Dans ce contexte, il nous paraît souhaitable de généraliser les meilleures pratiques afin de construire autour des jeunes de notre pays un environnement aussi sécurisant que possible. Nous sommes conscients qu'il faudra du temps pour mettre en place les procédures et les actions de formation et de sensibilisation adaptées, mais c'est le cap que nous nous sommes fixé et que nous vous proposons de suivre.

Je pense que le jeu des questions-réponses nous donnera l'occasion d'y revenir et d'explorer les autres mesures à mettre en oeuvre pour atteindre nos objectifs. Nous avons consacré une part importante de nos travaux aux infractions sexuelles commises au sein de l'Église catholique et au sein des autres cultes, ce qui était légitime compte tenu de l'actualité. Comme nous l'avons plusieurs fois entendu au cours de nos auditions, l'agression sexuelle commise par un religieux est particulièrement dévastatrice pour la victime, car à la violence physique et à la violence psychologique s'ajoute un abus spirituel qui peut être extrêmement déstabilisant. Nous avons perçu au sein de l'Église une prise de conscience réelle de la gravité du problème et une volonté affirmée de mettre un terme à l'omerta qui a longtemps prévalu. Nous avons tenté d'analyser les raisons de cette culture du secret, qui présente selon nous un caractère systémique, et nous avons rappelé l'absolue nécessité de signaler à la justice les faits délictueux ou criminels, en étant attentif à la parole des victimes, trop longtemps étouffée par peur du scandale. Nous avons pris acte de la volonté de l'Église d'indemniser les victimes, même pour des faits qui ne pourraient être jugés en raison de la prescription, ce qui nous paraît constituer une avancée importante. Nous devons rester vigilants afin de nous assurer que ces déclarations seront bien suivies d'effets. Nous formons le voeu que la commission Sauvé poursuive le travail visant à mettre au jour les infractions qui ont été commises et propose des mesures complémentaires.

Nous n'avons pas toujours perçu de la part des gestionnaires d'établissements et de services pour mineurs handicapés une prise de conscience de ce problème à la hauteur de la vulnérabilité du public qu'ils accueillent. Il nous semble que les contrôles effectués au moment du recrutement et la sensibilisation des professionnels qui travaillent auprès de ces mineurs pourraient être significativement renforcés. Les rapporteures et moi-même vous avons remis notre rapport au cours de l'été, monsieur le secrétaire d'État. Nous vous remercions de votre écoute, et je souhaite bien sûr que nos réflexions inspirent l'action du Gouvernement dans les prochains mois et les prochaines années. Le Gouvernement a récemment installé une commission pour les 1 000 premiers jours de l'enfant, qui devrait intégrer dans sa réflexion la prévention de la maltraitance. Je sais, monsieur le secrétaire d'État, que vous travaillez également sur le dossier de l'aide sociale à l'enfance et que vous préparez un plan de lutte contre les violences dont sont victimes les mineurs. Il prendra la suite du plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants 2017-2019 que notre collègue Laurence Rossignol avait mis en place lorsqu'elle était ministre chargée des familles. Peut-être pourrez-vous nous donner aujourd'hui de premières indications sur le contenu de ce plan. tout cas être assuré du soutien du Sénat à une politique ambitieuse de protection de l'enfance qui devrait constituer, à mes yeux, une grande cause nationale. Nos concitoyens attendent de notre part des décisions et des actes. Je ne doute pas que, sur un sujet comme celui-ci, un consensus pourra se dégager autour de quelques orientations fortes et d'un ensemble de mesures concrètes de nature à améliorer la protection des enfants et des adolescents dans notre pays. La parole

de la formation des professionnels, mais également celle de la prise en charge des auteurs- qui constitue souvent un angle mort de ces politiques. S'il ne règle pas à lui seul les insuffisances qu'il soulève, ce rapport d'information formule des propositions dans la recherche et la mise en place de solutions pour mettre fin aux violences en institutions.

au cours de nos échanges. Le sujet de vos travaux, plus largement la question de la lutte contre toutes formes de violences faites aux enfants, est au coeur de mes préoccupations. Le nouveau plan de lutte contre les violences faites aux enfants, que j'annoncerai prochainement, très probablement dans le courant du mois de novembre, à l'occasion du trentième anniversaire de

Nous pouvons donc travailler pour que cet observatoire nous permette d'appréhender de manière plus fine, plus précise, les violences sexuelles sur les mineurs, plus particulièrement dans les institutions, mais, à ce stade, et nous en rediscuterons, je ne suis pas sûr qu'il soit opportun de créer un nouvel outil. Appuyons-nous sur ce qui existe déjà. Concernant les chiffres dont nous disposons à ce jour, l'ONPE, vous le savez, publie chaque année un rapport comprenant, d'une part, des données chiffrées relatives aux mineurs pris en charge et, d'autre part, une analyse qualitative de l'évolution du dispositif de protection de l'enfance. Dans son dernier rapport, l'Observatoire a poursuivi sa collaboration avec le service statistique ministériel de la sécurité intérieure concernant la population des mineurs victimes de violences physiques et sexuelles. Les chiffres dont nous disposons, je l'ai dit, sont édifiants et nous obligent à faire mieux pour protéger nos enfants. En 2017, les forces de sécurité ont enregistré 22 000 mineurs victimes de violences sexuelles, soit un nombre en hausse de 10 % par rapport à Des enquêtes dites « de victimisation » montrent également qu'il existe un écart très important entre ce qui est porté à la connaissance des forces de sécurité et la réalité. Le taux de victimisation est à son plus haut niveau pour les mineurs de sexe féminin, puisque, en 2017, 2,5 mineures sur 1 000 ont déclaré avoir été victimes de violences sexuelles. Face à ce fléau, je ne pense pas que la meilleure piste soit de s'engager

Elle a également allongé le délai de prescription pour les personnes ayant subi des faits alors qu'elles étaient mineures. Il est important de rappeler ces

La méconnaissance des textes, conjuguée à une absence de lisibilité, conduit actuellement à un contrôle insuffisant par de nombreuses administrations. Il est indispensable d'engager une action forte pour coordonner et soutenir l'action des ministères afin de garantir une consultation plus systématique du

Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé.

En raison de leur grande vulnérabilité, les mineurs handicapés sont plus particulièrement exposés aux risques de subir des violences sexuelles en institutions. Par ailleurs, la multiplication des personnes intervenant auprès des mineurs handicapés augmente le risque d'agression. La mission d'information a tout particulièrement exprimé sa préoccupation sur le décalage qu'elle a perçu entre la vulnérabilité des mineurs handicapés et la faiblesse des contrôles effectués au moment du recrutement par les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui les accueillent. accueillent. Elle a également indiqué qu'elle n'avait pas non plus perçu chez les grandes associations qui fédèrent ces établissements et ces services une mobilisation à la hauteur des enjeux. Public fragile, vulnérable, exposé aux risques de subir des violences sexuelles tout en étant peu à même de les dénoncer, les mineurs handicapés doivent être mieux protégés, non seulement par une application stricte des contrôles exigés par la loi, mais également par des mesures supplémentaires. Ainsi, la mission d'information a fait part de la nécessité de renforcer les moyens de contrôle en mettant en oeuvre trois mesures : la diffusion par les services de l'État d'une information claire sur les procédures de contrôle à appliquer par les gestionnaires lors d'un recrutement

; l'application de ces mesures de contrôle aux employés des prestataires de services des établissements susceptibles d'être en contact avec des mineurs handicapés. Monsieur le secrétaire d'État, à la lumière des travaux de la mission d'information, quelles mesures envisagez-vous de prendre afin de mieux protéger les mineurs handicapés accueillis en institutions et dans quel délai ? La parole

Le rapport coordonné par M. Delarue a montré que ces insuffisances sont dues à la faible dénonciation des violences sexuelles par les victimes, à la proportion importante de plaintes classées sans suite et à l'extension de l'injonction de soins dans un contexte de pénurie de praticiens, vous l'avez évoqué. Un protocole santé-justice prévoit une coordination régionale des acteurs sur ce sujet. Au sein de chaque région, l'ARS et la direction interrégionale des services pénitentiaires mettent en place des protocoles locaux, qui fixent un projet d'organisation des soins et les modalités d'organisation matérielle de cette prise en charge. Ce protocole associe un établissement de santé chargé en général de la psychiatrie à chaque établissement pénitentiaire. Les centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles qui ont été créés en 2006 sont régionalisés de la même façon. Aujourd'hui vingt-cinq CRIAVS sont en fonctionnement sur l'ensemble du territoire et assurent un rôle de formation et de coordination. Ces centres sont aussi un lieu de soutien et de recours pour les équipes soignantes et participent de plus au développement et à l'animation du réseau santé-justice. Une action a été engagée ces dernières années pour renforcer la continuité de la prise en charge sanitaire des condamnés pour infractions sexuelles lors de leur sortie de détention. d'assurer une meilleure coordination entre les intervenants en milieu carcéral et ceux qui sont chargés du suivi du condamné en milieu ouvert. Cet objectif est partagé par la ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la justice. Il figure dans la feuille de route 2019-2022 pour la santé des personnes placées sous main de justice. Pour aller dans votre sens

Que fait-on quand un adulte sait déjà depuis longtemps qu'il est attiré sexuellement par de jeunes, tout jeunes enfants, ou de très jeunes adolescents ?

Une campagne nationale d'information, tant sur son numéro vert que sur la plateforme PedoHelp, est également préconisée. Ces initiatives me semblent fondamentales pour répondre aux difficultés des pédophiles avant que leur agression destructrice ne prenne une tournure pénale. Toutes

cours des dernières années, une association a incarné le combat mené pour dévoiler les agressions pédocriminelles graves et les porter sur la place publique. D'abord limitée aux violences sexuelles sur mineurs émanant du clergé catholique, cette parole poursuit sa libération partout ailleurs. Ma collègue Marie-Pierre de la Gontrie reviendra sur la genèse de notre rapport et sur ses conséquences dans l'Église. Pour ma part, j'évoquerai les pistes que nous traçons pour accueillir la libération de la parole, afin qu'elle ne soit pas vaine. Un enfant sur cinq est confronté à la violence sexuelle d'un adulte. Nous devons donc collectivement apprendre à nos enfants à parler des faits qui les dérangent dans leurs relations les adultes qui les entourent. Nous devons également apprendre aux adultes à écouter la parole des enfants. Ensuite, il faut signaler ces suspicions, sans hésitation. La plateforme du 119 doit être renforcée : nous demandons des campagnes de communication et de sensibilisation pour la faire davantage connaître. Quels moyens allez-vous y consacrer, monsieur le secrétaire d'État ?

faut faire évoluer les mentalités : il faut cesser de penser qu'on s'occuperait un peu trop de ce qui ne nous regarde pas. Pour cela, les professionnels et les bénévoles qui signalent ces violences doivent être informés des suites

Ce n'est pas possible. Nous allons donc développer, généraliser, pérenniser les UAMJP. Enfin, les cellules de recueil des informations préoccupantes, qui sont des maillons importants dans notre dispositif de signalement,

propositions auxquelles ont abouti nos échanges contribueront, si elles sont suivies d'effets, monsieur le secrétaire d'État, non seulement à briser ce tabou, mais aussi à mettre en oeuvre une politique globale de prévention de la pédocriminalité. Les propositions du rapport ne sont pas suffisantes à mes yeux en ce qui concerne la problématique, tabou des tabous, des violences sexuelles intrafamiliales envers les mineurs, autrement dit les violences à caractère incestueux, même si je sais que la mission ne traitait Si la loi votée en août 2018 a instauré un arsenal de mesures utiles et nécessaires, je regrette que, lors de l'examen de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, aucun de mes amendements proposer une surqualification pénale de l'inceste n'ait été repris par le Gouvernement. J'estime en effet qu'il est urgent de durcir la pénalisation des infractions sexuelles à caractère incestueux. Ce dossier doit être ouvert à la réflexion des parlementaires.

On estime que 6 % de la population américaine a été victime d'inceste. La seule étude, déclarative, qui a été faite en France conclut que 4 millions de nos concitoyens ont été victimes d'inceste,

Toutes les mesures que nous allons annoncer en novembre prochain auront aussi pour but

au sujet de la surqualification pénale de l'inceste. Bien sûr, dans le prolongement du rapport d'information dont nous débattons aujourd'hui, je salue la constitution par le Sénat du groupe de travail sur l'obligation de signalement des violences commises sur mineurs pour les professions tenues au secret. Je suis favorable à une telle mesure, que nous avions d'ailleurs demandée en vain lors de l'examen de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Nos recommandations, monsieur le secrétaire d'État, sont souvent qualifiées d'intéressantes,

a été signé entre le procureur et l'archevêque de Paris, et ce pour une période d'expérimentation d'un an. Cette démarche, déjà entreprise par les parquets avec d'autres institutions telles que l'éducation nationale ou les hôpitaux, est inédite pour l'Église. Elle va dans le bon sens : d'abord, parce qu'elle enclenche une dynamique de facilitation des signalements ; ensuite, parce qu'elle a le mérite de responsabiliser les parties prenantes. Cependant, ce genre de protocole nous interroge déjà par son caractère expérimental et coopératif. L'existence d'un tel dispositif met notamment au jour nos lacunes juridiques en matière de signalement des violences sexuelles sur mineurs. Certains acteurs auditionnés par la mission d'information ont en effet souligné que l'option de conscience permettant aux personnes soumises au secret professionnel de dénoncer des infractions sur mineurs ne suffit pas à établir un cadre légal lisible. Cette clarté constitue pourtant un enjeu primordial, à la fois pour protéger l'enfant victime de violences sexuelles et le professionnel susceptible d'en avoir connaissance. Le rapport d'information préconise d'ouvrir une réflexion sur l'introduction dans le code pénal d'une obligation de signalement pour les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les ministres du culte lorsqu'ils constatent qu'un mineur est victime de violences physiques, psychiques ou sexuelles.

dans le cadre de la stratégie nationale pour la protection de l'enfance, envisagez-vous de prendre des mesures pour garantir que les violences sur mineurs soient signalées ? La parole

226-14 du code pénal prévoit une levée du secret professionnel médical en cas de suspicion permettant de présumer des violences physiques, psychiques ou sexuelles. Les dispositions existantes sont cohérentes avec le caractère subsidiaire de l'intervention judiciaire par rapport à la protection de l'enfance, tant en termes de repérage que d'intervention. Dans ce cadre, introduire une obligation de signalement au sens judiciaire du terme serait contre-productif, et ce pour trois raisons. Premièrement, cela risquerait de mettre en péril la centralisation des informations à la CRIP, et donc sa capacité à évaluer correctement les situations. Deuxièmement, l'autorité judiciaire serait engorgée par des signalements, qui, par la suite, ne seraient pas évalués correctement ni croisés avec d'autres informations, mais simplement classés. Troisièmement, une telle obligation pourrait donner lieu à des placements judiciaires intempestifs, alors qu'une évaluation par la CRIP ou une intervention au niveau administratif aurait pu suffire. En revanche, nous souhaitons faire en sorte que l'obligation de transmettre des informations préoccupantes soit pleinement respectée par les professionnels. C'est le sens sous-jacent de votre question. Un travail prenant en compte deux difficultés que nous avons pu repérer est engagé : les professionnels ne sont pas suffisamment sensibilisés et informés, et les institutions ne font pas remonter les signalements en interne. Ainsi, un guide relatif à la prise en charge des mineurs victimes à destination des professionnels est en cours d'actualisation et devrait être prochainement diffusé à l'ensemble d'entre eux.

Dès l'enfance, ce sont des vies brisées. Dès lors, quelle est la réponse du Gouvernement à cette pandémie ? Quelle réponse l'exécutif souhaite-t-il donner à ces enfants souffrant de traumatismes durables ? C'est pour répondre à ces attentes que le Sénat s'est saisi de cette thématique par le biais d'une mission d'information. Par nos travaux, nous avons notamment constaté l'absence de moyens mis en place afin d'aider les victimes à surmonter leur psychotraumatisme manque de formation des praticiens médicaux, manque d'infrastructures spécialisées aux besoins psychiatriques et infantiles, prise en charge incomplète des frais médicaux. Le chemin est encore long pour que nous donnions aux victimes le suivi qu'elles méritent. Mes questions sont donc les suivantes dans un contexte où la psychiatrie des mineurs est sinistrée, quels moyens seront mis en place afin de mettre fin à ces déserts médicaux ? Enfin, prévoyez-vous la prise en charge intégrale des frais médicaux d'accompagnement psychologique ? La parole

pour la réplique. Vous n'avez pas répondu à ma deuxième question : prévoyez-vous la prise en charge intégrale des frais médicaux d'accompagnement

par sa présidente et les corapporteures. Le rapport formule des propositions utiles et pertinentes qui permettront d'avancer dans la prévention, la prise en charge des victimes, mais aussi des auteurs, ainsi que dans la connaissance du phénomène.

par la commission mixte paritaire. Une mission commune aux commissions des affaires sociales et des lois travaille actuellement sur cette question spécifique du signalement. Il me paraît en effet nécessaire de poursuivre les investigations sur ce sujet pour clarifier le droit applicable, parfois méconnu, et franchir une étape supplémentaire au bénéfice de la protection des enfants. Car le signalement ne saurait être associé à la délation contraire, il s'agit d'une responsabilité qui peut sauver des vies. Le secret médical est certes un principe cardinal du code de déontologie médicale, mais il ne saurait supplanter la protection de de l'enfant. Je rappelle, à ce titre, que 5 % seulement des enfants victimes de violence sont détectés par les médecins. Ce chiffre est forcément trop faible. Par ailleurs, le nombre de médecins scolaires a chuté de 25 % ces dix dernières années.

Les textes existent, madame la sénatrice. Une obligation de dénoncer s'impose, y compris au dépositaire d'un secret professionnel lorsque le crime ou le délit est susceptible de se produire. Si une meilleure connaissance de la procédure de signalement par les praticiens de santé apparaît nécessaire, des outils existent et un travail est engagé pour améliorer leur diffusion, je l'évoquais précédemment. La systématisation d'une obligation de signalement pour l'ensemble des infractions pénales pourrait avoir pour conséquence d'entamer la confiance dont bénéficient au premier chef les professionnels de santé et d'empêcher le recueil d'informations préoccupantes, ou encore de constituer un obstacle supplémentaire aux soins nécessaires aux enfants victimes, sans compter le risque de noyer les services départementaux. En réalité, le problème ne

Ainsi, au sein des établissements d'accueil du jeune enfant agréés par les conseils départementaux et dans ceux agissant dans le cadre de la protection de l'enfance, seul le bulletin n° 2 du casier judiciaire est interrogé. Il en va de même pour le contrôle effectué pour les employés travaillant au contact des enfants handicapés. C'est aussi le cas lors de la procédure d'agrément des assistantes maternelles par les services du conseil départemental. Ce contrôle paraît largement insuffisant au regard de la vulnérabilité des publics concernés. Mais, plus encore, il arrive que ces structures, pour faire face à des absences ou a un manque de personnel, soient contraintes d'embaucher à titre temporaire du personnel moins qualifié, parfois même sans diplôme. Elles n'interrogent alors que très rarement le bulletin n° 2, et le président du conseil départemental ne peut exercer son contrôle sur les recrutements. comment rendre obligatoire par les organismes employeurs la consultation du FIJAISV avant tout recrutement, quel qu'il soit ?

se décompose en trois sous-questions : les conditions d'inscription à ce fichier, les conditions de consultation et les modalités de mise en oeuvre de cette consultation auxquelles sont confrontées un certain nombre de collectivités ou d'associations.

conformes à la réalité de l'activité des personnes concernées. C'est ce que nous devons développer. En partenariat étroit avec le ministère de la justice, nous travaillons ainsi à garantir, par une action interministérielle d'envergure,

Au-delà de l'évolution normative et technique, nous devons mener une réflexion quant à la société que nous voulons pour nos concitoyens et leurs enfants. C'est un sujet sensible qui allie la protection des mineurs, mais aussi la liberté individuelle et la protection des données. Je vous invite à conclure ! Pour moi, la protection des mineurs est supérieure à toute autre chose.

de Mme Bachelot et de. En quelques jours, 30 000 signatures ont été recueillies. Le Sénat, pour des raisons qui lui appartiennent, a refusé la création de cette commission d'enquête, et la mission d'information est née. Vous l'avez dit, tous les citoyens doivent se mobiliser.

Aux États-Unis, un procureur de Pennsylvanie a identifié 300 prêtres pédophiles. En Belgique, une commission parlementaire a été mise en place. En France, c'est la Conférence des évêques qui a créé la commission Sauvé,

Que fait l'État face à cela ? Je ne me prononcerai pas sur la décision qui a été prise par cette noble assemblée ; cela ne relève pas de l'exécutif.

même si la victime n'a pas porté plainte, de façon dérogatoire. Cela contribue à libérer la parole et à éviter que des affaires restent enfouies ou non traitées. En outre, vous l'avez dit, la commission indépendante présidée par Jean-Marc Sauvé est chargée d'enquêter sur les abus sexuels commis sur les mineurs depuis les années cinquante. Elle bénéficie du soutien de l'État, de l'Inserm, qui analysera les témoignages, de la Maison des sciences de l'homme, qui produira des monographies sur des congrégations et diocèses déterminés,

est à Mme Chantal Deseyne. Ma question porte sur l'évaluation de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dite loi Schiappa. Si cette loi a permis plusieurs avancées pour protéger les mineurs contre les infractions sexuelles, elle est loin d'avoir répondu à toutes les attentes, notamment des associations de victimes. Il suffit d'analyser les décisions judiciaires prises depuis l'entrée en vigueur de la loi pour comprendre que les jugements ne sont toujours pas à la hauteur des enjeux. Je ne citerai que l'affaire du Mans concernant ce grand-père récidiviste ayant commis un viol sur sa petite-fille âgée de huit ans. Alors qu'il encourait théoriquement vingt ans de réclusion pour viol devant une cour pour viol devant une cour d'assises, il a été condamné, en mars dernier, par un tribunal correctionnel, à huit mois seulement, et avec sursis ! Beaucoup d'experts doutent que la loi suffise à mettre fin à la correctionnalisation des procédures, au détriment des victimes. Près de quinze mois après son entrée en vigueur, il est donc souhaitable d'en évaluer les effets, un souhait d'ailleurs partagé par le Gouvernement, monsieur le secrétaire d'État, puisque vous avez récemment confié une mission d'évaluation à la députée Alexandra Louis. Alexandra Louis. Ma question est double. Premièrement, la garde des sceaux Nicole Belloubet a déclaré en juin dernier à l'Assemblée nationale que la loi Schiappa contenait des évolutions positives dont les juges s'étaient déjà emparés. Pouvez-vous nous faire part de vos premiers retours d'expérience permettant de mesurer l'impact de cette loi ? Conduit-elle les juges à retenir plus fréquemment la qualification de viol ? Permet-elle aux victimes déposant plainte plus de trente ans après les faits de faire condamner plus facilement leur agresseur ou aboutit-elle au contraire à des classements sans suite décevants ? Ma deuxième question a davantage trait à la méthode que vous avez choisie pour procéder à l'évaluation de la loi. Accepteriez-vous de confier cette démarche d'évaluation à un collège pluraliste associant députés et sénateurs ?

Tous les mois, la presse se fait l'écho de scandales insupportables au sein même des institutions qui accueillent des enfants et qui ont aussi pour mission de les protéger. Ainsi, le 23 septembre dernier, au Mans, une éducatrice a été condamnée pour des atteintes sexuelles sur mineurs commises entre 2011 et 2018. Deux jours plus tard,

Comment est-il possible que des personnes condamnées pour exhibition sexuelle puissent encore travailler au sein d'institutions accueillant des enfants ? Le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, le FIJAISV, a justement pour objectif de prévenir la récidive des personnes déjà condamnées.

En partenariat étroit avec la garde des sceaux, nous travaillons à essayer de garantir que l'arsenal législatif dont nous disposons soit effectivement appliqué. effectivement appliqué. Nous devons pour cela évaluer la mise en oeuvre des dispositions récentes de la loi du 14 avril 2016 et mieux appréhender les difficultés rencontrées, pour rendre le cas échéant cette obligation plus effective.

De nombreux sportifs ont récemment fait état de tels comportements à leur égard. Cette prise de conscience est importante, même si elle est encore trop faible. Leur mobilisation, comme celle, croissante, des pouvoirs publics, est une réelle avancée que nous devons profondément encourager. La difficulté que le monde sportif rencontre pour lutter contre les violences sexuelles tient à l'absence de données sur le nombre d'actes et l'âge des victimes. Mais elle vient aussi d'un manque d'information et d'une véritable omerta sur le sujet. Trop souvent, les enfants se murent dans le silence. L'association Colosse aux pieds d'argile, reconnue pour ses engagements contre les violences sexuelles dans le milieu du sport, nous rappelle que ces violences toucheraient environ 10 % des sportifs et 13 % des sportives. Lors des auditions de notre mission, il a été souligné que la majorité des violences sexuelles commises dans le sport sont commises entre sportifs. Il n'en Il n'en demeure pas moins qu'il existe malheureusement trop d'abus sexuels commis sur des enfants par un éducateur sportif ou un entraîneur. Je rappelle que, depuis 2015, près d'une centaine de cas d'éducateurs inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ont été recensés. De nombreux trous dans la raquette demeurent toutefois. Aussi, monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous informer des mesures que compte prendre le Gouvernement sur la formation et l'information des éducateurs sportifs et des entraîneurs, mais aussi des présidents d'association, pour mieux les sensibiliser et les accompagner dans leurs missions ? leurs missions ? La ministre des sports avait annoncé vouloir expérimenter un dispositif de contrôle des casiers judiciaires des bénévoles, afin de protéger les jeunes licenciés. Qu'en est-il ?

par quel biais pouvons-nous contrôler l'honorabilité des bénévoles ? Faut-il en passer par une licence ou un autre dispositif ? La ministre est en train d'expertiser

plaintes pour viol et 14 673 plaintes pour atteintes sexuelles sur mineurs ont été enregistrées. Mais combien de souffrances échappent à notre lecture ? Comme le disait le juriste Denys de Béchillon, la correction des erreurs doit pouvoir suivre l'essai ; l'auteur de la norme doit pouvoir la reprendre ou l'amender assez aisément si l'expérience l'a vérifiée inappropriée, inefficace, voire dangereuse. Ainsi, une double prévention est nécessaire le signalement par l'entourage, d'une part, la facilitation de la libération de la parole, d'autre part. En complément, un recueil d'informations plus large doit également être établi. En effet, les démarches visant à accroître la connaissance du phénomène sont consubstantielles à celles qui visent à l'enrayer. Ces démarches doivent avoir pour triple finalité de déterminer selon quels indicateurs évaluer l'efficacité des mesures, vers quels secteurs porter l'attention du législateur et quelles sont les méthodes de prévention ou de lutte contre la récidive les plus appropriées dans les institutions. Je tiens à saluer l'excellent et Je tiens à saluer l'excellent et remarquable travail réalisé par la mission commune d'information, en particulier par sa présidente, Catherine Deroche, ainsi que par nos collègues Marie Mercier, Michelle Meunier et Dominique Vérien, dont le rapport propose la création d'un observatoire national des violences sexuelles sur mineurs, affilié à l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Cet observatoire aurait notamment pour rôle la réalisation d'enquêtes épidémiologiques et criminologiques, sur le modèle de l'enquête Virage sur les violences faites aux femmes. Cette enquête aurait évidemment

de l'enfance. Comme vous le savez, elle est partagée entre l'État et les départements, qui en assurent la mise en oeuvre très concrète dans les territoires. Nous devons améliorer

Stéphane Piednoir. La mission d'information du Sénat ne traitait pas des infractions sexuelles commises dans le cadre familial, mais nous savons, chiffres à l'appui, que ce sont de loin les plus nombreuses. L'un des axes de nos travaux porte en revanche sur la prévention de ces actes. Or, après les membres de la famille, les enseignants sont les adultes les plus fréquemment en contact avec les enfants et adolescents. Ils ont donc, de fait, un rôle non négligeable à jouer dans la détection des infractions sexuelles qui pourraient être commises à l'encontre de leurs élèves. Sans prétention d'exhaustivité, nos auditions ont permis de dégager des « signaux d'alerte » qui peuvent permettre de reconnaître un enfant ou un adolescent victime : : changement brutal de comportement ou de niveau scolaire, apparition de troubles auparavant absents, gestes sexualisés sans rapport avec ce qui est habituel pour un enfant de cet âge, etc. Aussi, pour que davantage d'infractions sexuelles puissent être détectées et ainsi stoppées dès le plus jeune âge, il me paraît essentiel d'intégrer à la formation des enseignants de l'éducation nationale un volet lié à l'identification de ces signes.

Or nous avons constaté que l'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire n'est souvent pas effective, alors qu'elle pourrait justement permettre aux jeunes d'identifier plus facilement les limites que les adultes ne doivent pas franchir dans le cadre d'une classe. Là encore, les enseignants sont souvent peu formés et incapables de dispenser de tels « enseignements » à leurs élèves. Monsieur le secrétaire d'État, j'en suis convaincu, la formation et la sensibilisation des

Ils sont dans une position privilégiée pour transmettre les valeurs de respect du corps et de la dignité, sensibiliser les enfants aux violences sexuelles et repérer les situations d'abus ou de maltraitance. Il est donc essentiel qu'ils soient formés aux comportements à adopter, aux informations à communiquer et aux procédures à mettre en oeuvre.

pour le personnel scolaire. Dans le cadre de la formation continue, l'accent est mis sur la sensibilisation au repérage de signaux d'alerte, la connaissance du fonctionnement des dispositifs départementaux ou encore l'acquisition de compétences pour protéger les enfants en danger ou qui sont susceptibles de l'être.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat, organisé à la demande de la commission des affaires sociales, sur la santé en Guyane. Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses, dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ce vaste territoire de France couvert de forêt amazonienne qu'est la Guyane possède, nous le savons tous, d'innombrables atouts pour des raisons évidentes, tenant à sa géographie et également du fait de son contexte démographique et social, la Guyane fait aussi face à des défis singuliers.

plaquer la même grille de lecture sur tous les territoires serait évidemment inopérant. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que le Sénat consacre un temps spécifique à la santé en Guyane. Je me réjouis donc de la tenue de ce débat, qui nous permet de faire le point sur l'action menée par le Gouvernement, plus de deux ans après les accords de Cayenne, qui ont mis fin à un mouvement social dans lequel les questions de santé étaient sous-jacentes.

La démographie, cinq fois plus dynamique que la moyenne nationale, met tout le système en tension. Nous avons rencontré des équipes de soins engagées et dévouées, à l'instar de celles de métropole, mais que leur environnement général conduit, en pratique quotidienne, à l'épuisement

Cette crise prend racine dans des déterminants multiples et profonds. L'accès aux soins figure au premier rang de ces défis. des zones de l'intérieur le transforme en parcours du combattant pour une partie de la population. De fait, moins de la moitié des dix-huit centres délocalisés de prévention et de soins qui maillent le territoire offrent une présence médicale continue. Dans ce contexte, des initiatives intéressantes nous sont apparues encore trop peu exploitées, comme le développement d'hôtels hospitaliers permettant de réduire la pression sur les services.

Sans surprise, l'ensemble de la Guyane est classé déficitaire en offre de soins, avec moins de 600 médecins en activité. L'hôpital subit les carences de l'amont- l'offre libérale parfois quasi inexistante -comme de l'aval- des structures médico-sociales d'accueil en nombre largement insuffisant. Tous les métiers de la santé sont en souffrance, fait, dans certaines spécialités, particulièrement criant. C'est le cas en pédiatrie et en néonatalité, alors que la Guyane enregistre 9 000 naissances par an et que 40 % de sa population a moins de vingt ans. Bien évidemment, en Guyane comme dans toutes les régions, la question de l'attractivité pour les professionnels de santé est étroitement corrélée à des enjeux plus globaux d'attractivité du territoire, auxquels les élus guyanais sont particulièrement attentifs. que des leviers d'action sont mobilisables pour adapter l'organisation de l'offre de soins à ces défis. Ainsi, il me semble que la Guyane devrait être à l'avant-garde de la transformation souhaitée de notre système de santé, en s'appuyant sur l'innovation.

Les enjeux de la formation des professionnels de santé sont également majeurs. J'appelle votre attention, monsieur le secrétaire d'État, sur l'importance d'offrir sur place des terrains de stage aux futurs médecins et de développer les formations d'infirmier et de sage-femme. Sans être un CHU, le centre hospitalier de Cayenne présente des services de pointe, par exemple en matière de maladies infectieuses, qui méritent de servir de centres de référence au plan national et de catalyseurs de l'attractivité médicale dans la région. Il me semble également que nous ne tirons pas pleinement parti du recours, déjà possible en Guyane, à des médecins diplômés hors de l'Union européenne ; la réflexion nous a souvent été faite, monsieur le secrétaire d'État, et je crois qu'il faut en tenir compte.

intransigeants sur la qualité de la formation de ces médecins. Nous pensons en particulier à Cuba, où la formation à la médecine est particulièrement intéressante. Alors que le Gouvernement a missionné sur place de multiples experts, pouvez-vous nous éclairer, monsieur le secrétaire d'État, sur les leviers que vous entendez actionner pour répondre à l'urgence de l'attractivité médicale de la Guyane et au malaise de ses équipes de soins ? rejoignent pour partie la situation exceptionnelle de Mayotte, où j'ai souhaité que la commission se rende en mission l'année la pression migratoire accentue les enjeux d'accès aux droits et aux soins. Pour ces deux territoires, le Premier ministre a confié en 2018 à notre ancienne collègue Dominique Voynet et au préfet Marcel Renouf une mission sur la coopération transfrontalière. Quelles

Aucune question ne trouve de réponse aisée, mais vous pouvez compter, monsieur le secrétaire d'État, sur notre volonté partagée de rechercher ensemble les solutions les mieux adaptées aux défis sanitaires d'un territoire riche de sa jeunesse et de sa diversité.

Il avait compris bien avant nous la richesse de ce territoire, ses spécificités et ses défis, immenses, à la mesure

25 millions d'euros ont été attribués dès 2017 au centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Maroni pour lui permettre de faire face à son budget d'investissement. Le centre médico-chirurgical de Kourou, mis en vente par la Croix-Rouge, a été transformé en hôpital public. l'hôpital de Cayenne, il a bénéficié d'un abondement exceptionnel de trésorerie de 20 millions d'euros, ainsi que de 40 millions d'euros pour un programme spécial d'investissement. Au-delà de la nécessité de s'atteler à la rénovation des infrastructures,

La densité de médecins généralistes libéraux est en Guyane plus de deux fois inférieure à celle observée dans l'Hexagone, et les autres professions de santé sont également caractérisées par des effectifs et des densités pour 100 000 habitants très faibles relativement à d'autres territoires, et de manière générale à l'Hexagone.

dans le cadre du comité interministériel de la santé, le Premier ministre et la ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, ont présenté les mesures du plan Priorité prévention, parmi lesquelles figure la création, sur des crédits de l'assurance maladie, de 100 postes d'assistant spécialiste à temps partagé avec une obligation d'exercice en outre-mer, par recrutement annuel de 50 postes, à partir de novembre 2018. Cette mesure répond au double objectif de renforcer l'offre locale de soins et de participer à la réduction des inégalités territoriales, inscrit dans la stratégie nationale de santé et que nous déclinons spécifiquement pour l'outre-mer. Enfin, l'ARS de Guyane a conclu une convention avec l'AP-HP aux fins de

pour pouvoir recevoir des citoyens de ces pays limitrophes quand cela est nécessaire, tout en contrôlant l'afflux de ces femmes et de ces hommes qui, parfois, peuvent empêcher l'accès aux soins ou le rendre plus difficile encore.

Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé.

La pédiatrie, la protection maternelle et infantile, le handicap, le nombre de places en Ehpad : autant d'indicateurs qui virent au rouge, alors que nous parlons de l'accompagnement d'un public vulnérable sur un territoire, vous

Entre 2016 et 2018, environ 50 millions d'euros d'aides exceptionnelles ont été versés à l'établissement, tandis que 9 millions d'euros ont été accordés en revalorisation pérenne de dotations. Les difficultés financières et la fragilité de l'équipe de direction ont conduit l'ARS à placer l'établissement sous administration provisoire entre novembre 2018 et avril 2019. Cette mission a permis notamment de conforter le schéma directeur immobilier, financé par l'État à hauteur de 40 millions d'euros, de travailler au renforcement de l'attractivité de l'établissement et de faire aboutir favorablement la démarche de certification des comptes, après plusieurs années de non-certification. Le centre hospitalier ouest-guyanais est également dans une situation de déséquilibre financier, mais sa reconstruction, qui a bénéficié d'une aide nationale de 48 millions d'euros,

pour mieux accompagner les patients et leur famille, lorsque la situation médicale l'exige.

pour traiter les patients sur place et former les équipes locales ; cette coopération permettra à l'équipe guyanaise de gagner en compétences et en autonomie, pour, à moyen terme, prendre en charge elle-même ses patients, y compris en urgence. Les patients les plus complexes continueront d'être pris en charge en Martinique, dans des conditions plus favorables, puisque les équipes auront appris à travailler ensemble. C'est donc un modèle de coopération gagnant-gagnant que nous souhaitons mettre en place et que la Guyane pourra dupliquer à d'autres filières de soins. Il s'agit, je le répète, de renforcer l'offre de soins sur place pour limiter les évacuations sanitaires, très lourdes à supporter pour les patients et leur famille.

Première étape dans la structuration de l'offre de soins hospitalière, ce regroupement est censé aider les centres hospitaliers de Saint-Laurent-du-Maroni, de Kourou et de Cayenne à mieux travailler ensemble, au bénéfice des patients.

Système de soins sous tension, désertification médicale, difficultés d'accès aux soins, formation des professionnels ... Mes collègues de la commission des affaires sociales ont pu l'observer : la Guyane doit relever de nombreux défis, amplifiés par le retard accumulé en matière d'infrastructures médicales.

ailleurs, le code de la santé publique prévoit que tous les groupements hospitaliers de territoire soient associés à un centre hospitalier universitaire. Pour l'heure, une de développement et d'attractivité. Je rappelle que la création d'un CHU en Guyane figure parmi les engagements du protocole d'accord du 9 juin 2017, arraché après soixante-quinze jours de grève et dont je suis l'un des cosignataires.

Contrairement aux craintes qui s'étaient exprimées avant sa constitution, le GHT prend forme. Les équipes médico-soignantes se voient régulièrement et travaillent sur un projet médical partagé. Une prochaine session est d'ailleurs prévue en octobre prochain à Sinnamary. Les hôpitaux s'entraident sur le plan de leurs ressources médicales par des envois réciproques de renforts ponctuels en fonction des besoins ; ils s'entraident aussi en orientant les patients entre eux. Ils travaillent sur une stratégie commune en matière de systèmes d'information, ainsi que de ressources humaines. Il s'agit, pour les hôpitaux publics, d'avancer de concert et de ne pas se faire de concurrence,

des trois établissements de santé, et ainsi contribuer à améliorer l'offre de soins sur le territoire. Les spécificités de chaque hôpital et de chaque territoire me semblent être mieux comprises et respectées. Soyez convaincu, monsieur le sénateur, de la forte volonté de l'agence régionale de santé de s'inscrire dans ce mouvement

Lors de ce déplacement, nous avons pu constater, outre les conséquences désastreuses de l'incendie du CHU de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, l'attente des Guyanaises et des Guyanais à la suite notamment du mouvement social de 2017, qui avait débouché sur les accords de Cayenne.

pourquoi un territoire tel que celui de la Guyane, qui compte près de 300 000 habitantes et habitants, ne dispose pas d'un centre hospitalier universitaire. En l'absence d'un CHU, les étudiantes et les étudiants guyanais sont contraints de quitter leur territoire pour terminer leur formation.

prérogative de l'université, qui dispose de sa propre stratégie de développement en tant qu'établissement autonome. Le développement de départements universitaires repose sur la définition d'une stratégie et la création de filières

Le programme « bien-être des populations de l'intérieur », doté de 1,5 million d'euros à débloquer sur trois ans, a été conçu avec la population pour soutenir l'émergence de projets locaux et renforcer les facteurs protecteurs, notamment liés à l'estime de soi. Sachez que l'ARS travaille en ce moment sur la mise en place de la formation nationale de prévention du suicide,

Les difficultés que nous connaissons en métropole sont exacerbées dans ce territoire et se surajoutent aux problématiques locales qui mettent déjà le système de santé sous tension. Les assises des outre-mer ont révélé que l'accès aux soins est la priorité absolue en matière de santé pour les Guyanais. La Guyane est à la fois le deuxième plus vaste territoire de France et le deuxième moins densément peuplé. Quelque 20 % de la population est issue de l'immigration, souvent clandestine, et ne dispose de ce fait d'aucune couverture sociale. Le taux de pauvreté de l'ensemble du pays atteint 44 %, et atteint 44 %, et le taux de fécondité 3,5 enfants par femme. L'éloignement de toute une partie de la population du système de santé retarde le dépistage, en particulier pour le VIH. présente une surmortalité liée au sida par rapport à la métropole. Les hôpitaux des villes frontalières telles que Saint-Laurent-du-Maroni sont particulièrement sollicités. Cela invite la France à développer des accords de coopération transfrontalière en matière de santé avec le Brésil et le Suriname. Au regard de la situation sociale et géographique de la Guyane, la politique sanitaire locale ne peut être une déclinaison de la politique sanitaire nationale. Nous devons l'adapter pour qu'elle réponde aux besoins de la population, comme le prévoit l'article 73 de notre Constitution. Monsieur le secrétaire d'État, les accords du 21 avril 2017 signés à Cayenne ont permis de débloquer un milliard d'euros, notamment pour venir en aide au système de santé du pays, qui peine à se moderniser.

une situation épidémiologique inquiétante et des populations isolées. Le Gouvernement, au travers des accords de Cayenne, a effectivement décidé d'investir massivement.

En tant que médecin, j'ai pu y constater un certain nombre de difficultés. Je n'imaginais pas qu'un territoire français puisse connaître des problèmes de santé que l'on ne voit

pour notre système de santé, en s'appuyant sur la créativité volontariste des équipes de terrain. Monsieur le secrétaire d'État, comptez-vous faire de la Guyane une zone prioritaire pour la mise en place d'expérimentations ? L'article 51

La Guyane s'est très vite mobilisée pour tirer parti de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018. Sur l'initiative des acteurs locaux et de l'ARS,

matière d'ophtalmologie, les équipes de l'ARS ont accompagné le centre hospitalier de Cayenne et un cabinet d'ophtalmologie de ville pour permettre la réalisation de petits actes chirurgicaux hors milieu hospitalier dans un cadre sécurisé et respectueux des conditions d'hygiène, incluant les patients dans une logique de filière ville-hôpital

villes-centres, Nouméa ou Cayenne, même si, en Calédonie, le territoire est mieux irrigué par des dispensaires et des maisons de santé, un hôpital ayant récemment été construit au nord. Parmi les points communs, je m'attarderai sur les difficultés des centres de santé, hôpitaux ou dispensaires à trouver des médecins, notamment spécialistes. Cette pénurie de médecins a des causes multiples que l'on connaît bien : le, la faible attractivité du statut des praticiens, notamment en ce qui concerne la rémunération, les contraintes de la profession en termes de garde la nuit et le week-end. En conséquence, non seulement nos territoires n'arrivent plus à attirer de médecins, mais en plus la sous-densité médicale conduit les médecins en place à l'épuisement,

du pays. Monsieur le secrétaire d'État, l'AP-HP a engagé un partenariat en 2018 avec la Guyane pour envoyer des médecins spécialistes dans les établissements déficitaires : où en est-on de ce partenariat ?

Guyane. En 2019, l'ARS de Guyane a mené une opération de promotion très offensive qui a permis de faire mieux connaître ce dispositif. L'évaluation finale de cette opération est en cours de réalisation. Par ailleurs, l'ARS de Guyane développe actuellement, en partenariat avec la caisse générale de sécurité sociale du territoire, une plateforme d'appui aux professionnels de santé permettant d'apporter des réponses claires, complètes et validées à tous les candidats potentiels et aux professionnels installés.

Elle facilite en effet l'intégration en Guyane de jeunes professionnels dont beaucoup craignaient une forme de solitude médicale. Pour accroître le déploiement de cette convention, convention, l'ARS de Guyane a recruté un agent de liaison entre la Guyane et l'AP-HP qui aide concrètement les professionnels à entrer en contact, à développer des projets de collaboration et à assurer leur pérennisation, bref à donner de l'ampleur au dispositif que nous avons créé. Enfin, concernant l'évolution des pratiques autorisées au personnel paramédical pour suppléer l'absence de médecins, le recours

La définition d'une politique de coopération sanitaire entre le Suriname et la Guyane viendrait non seulement organiser les rapports qui existent déjà, mais permettrait aussi de rééquilibrer la prise en charge des patients en tirant profit des atouts de chacune des structures hospitalières de part et d'autre du Maroni. De fait, les deux territoires ont en commun de devoir faire face à une situation sociale marquée par une grande précarité et un accès limité aux soins. Mais en Guyane, les conditions de prise en charge sociale relativement plus favorables génèrent une pression migratoire qui vient fortement grever les capacités d'accueil du centre hospitalier de l'Ouest guyanais. Ce nouvel établissement, que vous venez d'inaugurer, subit ainsi les mêmes contraintes que le précédent, à savoir une demande supérieure à sa capacité d'accueil, une patientèle souvent en situation irrégulière, voire ne parlant pas français. Or le fleuve Maroni, s'il matérialise une frontière, est aussi l'axe d'un bassin de vie qui pourrait constituer une zone de coopération sanitaire, voire un espace dans lequel un parcours de soins est envisageable. À cet égard, le Premier ministre avait souhaité qu'une étape significative de la redéfinition de la coopération sanitaire puisse être franchie avant septembre 2018 et confié une mission en ce sens à Mme Dominique Voynet. Pouvez-vous nous indiquer, monsieur le secrétaire d'État, quelles sont les pistes dégagées par cette mission et leur degré de mise en oeuvre ?

à Dominique Voynet et au préfet Renouf afin de renouveler les modalités de la coopération sanitaire entre la Guyane et le Suriname, mais aussi entre Mayotte et les Comores. L'objectif de cette mission était d'aboutir à la signature d'un accord entre les deux États qui aurait comporté un volet sanitaire substantiel.

Le dernier déplacement de la mission au Suriname a eu lieu entre les 3 et 6 avril dernier, pour une réunion du groupe de travail franco-surinamien sur la coopération en matière de santé. En parallèle de la mission, l'ARS a poursuivi ses travaux avec les autorités sanitaires du Suriname. Engagés depuis plusieurs années, ils ont pour objectif de rapprocher les communautés médicales des deux pays et d'accentuer la coopération selon les complémentarités des deux systèmes de santé. Une déclaration d'intention a été rédigée entre l'ARS et le ministère de la santé du Suriname en janvier 2017,

Ce qui est valable pour la Guyane l'est aussi pour les autres territoires et collectivités d'outre-mer. Une telle approche intégrée me semble être la meilleure des voies pour nos territoires et pour la France, mais elle nécessite, comme c'est souvent le cas, des solutions dérogatoires et innovantes

manque cruellement de moyens humains, au niveau tant médical que médico-technique, ainsi que d'équipements performants et adaptés à une pratique médicale et paramédicale de haute qualité.

Interrompues depuis 2005, les collectes de sang doivent reprendre de manière urgente. En effet, il est impératif de prélever le sang en Guyane pour répondre aux besoins de prise en charge des patients drépanocytaires,

des établissements guyanais à développer un projet médical se heurte à la situation de spécialités qui évolue « au fil de l'eau », au gré des arrivées et des départs de médecins. Certaines spécialités sont en souffrance de manière ponctuelle,

comptez-vous déployer pour renforcer le pôle hospitalier guyanais dans le respect des équilibres du territoire ? En l'absence de CHU, comment entendez-vous valoriser l'attractivité médicale et préserver les filières d'excellence sur ce territoire ?

établissement de référence, avec des activités d'excellence dans certaines disciplines médicales, en lien avec l'UFR de médecine de Guadeloupe. La création d'un CHU, une fois encore, est pour l'instant difficile à envisager.

et connaît une croissance démographique très forte. Ainsi, l'inégale répartition de l'offre de soins a pour conséquence une crise sanitaire qui s'accompagne indéniablement d'une grande précarité, d'autant que la Guyane est confrontée à de nombreuses pathologies infectieuses et chroniques ou à des problèmes spécifiques, comme la drépanocytose. Contrairement à ce qu'affirment certains, ce n'est pas à la Guyane de s'adapter au système de santé hexagonal, mais plutôt au système de santé de s'adapter à la Guyane Les Guyanais ne peuvent plus se contenter de trois hôpitaux et de dix-huit centres délocalisés de prévention et de soins dans des zones reculées et difficiles d'accès. L'offre de soins y est marquée par un niveau d'équipement de deux à trois fois inférieur à celui observé dans l'Hexagone ! Les projections démontrent en outre

que dire des forts besoins en matière de périnatalité, du retard important dans l'accueil des adultes handicapés, des difficultés rencontrées par les jeunes en insertion pour se procurer les médicaments qui leur ont été prescrits ? Il est plus que temps de mettre fin à cette crise permanente de l'offre de soins, car l'aide financière apportée par l'État n'effacera pas durablement le passif des hôpitaux de Cayenne, de Saint-Laurent-du-Maroni et de Kourou. Il faut des mesures d'urgence fortes et spécifiques. Cela pourrait passer par la création d'un nouveau CHU- cela est le développement d'une coopération régionale pérenne et l'annulation de la dette des hôpitaux publics. Monsieur le secrétaire d'État, envisagez-vous la mise en oeuvre de ces mesures d'urgence ? Quelles dispositions concrètes le Gouvernement entend-il adopter pour remédier à cette situation catastrophique ? La Guyane est une terre de paradoxes, terre des infinis : infiniment grande par sa capacité à permettre l'exploitation de l'espace, infiniment petite par son incapacité à lutter avec efficacité contre les petits virus pathogènes.

La création d'un CHU ne serait en rien une solution pour améliorer la prise en charge des Guyanais à Cayenne. Le recrutement de professionnels et d'une équipe de direction stable est un signe encourageant de redressement, nous semble-t-il. En outre, nous souhaitons travailler de concert avec la collectivité territoriale de Guyane pour renforcer les moyens de

Mme Chantal Deseyne. Monsieur le secrétaire d'État, notre commission a adopté au début du mois de juillet dernier un rapport formulant plusieurs propositions en vue de renforcer la prévention des infections par le VIH et d'améliorer la prise en charge des personnes vivant avec ce L'enquête que notre commission avait demandée à la Cour des comptes fait état d'une concentration des nouvelles infections dans trois régions : Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Guyane.

La situation est beaucoup plus problématique en Guyane, où l'accès aux traitements préventifs est nettement moins aisé. Pourtant, selon le comité de coordination

bien connu dans les domaines sanitaire et médico-social, avec des équipes mobiles de santé associées à des médiateurs culturels. La stratégie de prise en charge évolue progressivement vers une autonomisation des patients.

d'Oiapoque. Enfin, l'expérimentation « Au labo sans ordonnance » porte sur le remboursement d'un examen de biologie médicale non prescrit, réalisé à la demande du patient. Il s'agit d'un remboursement dérogatoire qui a été accepté jusqu'à présent par deux caisses primaires d'assurance maladie volontaires, celles de Nice et

criante par nos concitoyens ; nous l'avons encore constaté à l'occasion des mouvements sociaux de l'automne dernier. Il faut évidemment agir sur différents leviers : vous avez évoqué le réseau routier,